le Sénat a le devoir d'accomplir de manière adaptée sa mission constitutionnelle de contrôle de l'action du Gouvernement. Nous devons assurer la continuité de la vie démocratique de notre pays. Une autre séance de questions se tiendra la semaine prochaine. Je voudrais rappeler à nos compatriotes qui suivent nos débats l'importance du respect des mesures de confinement telles que demandées par le Gouvernement et qui sont fixées par la loi d'urgence sanitaire.

Avant de laisser la parole aux auteurs des questions, je voudrais vous faire part des suites données à nos débats de la semaine dernière sur le projet de loi d'urgence et sur le projet de loi de finances rectificative. Je vous ai adressé deux lettres, monsieur le Premier ministre, pour rappeler les engagements pris par le Gouvernement devant notre assemblée. Je souhaite en indiquer la teneur à nos collègues. La première rappelle que l'adoption sans modification du projet de loi de finances rectificative est, à la fois, une marque de confiance et d'exigence. Il reviendra au Gouvernement de travailler à l'élaboration d'une mesure simple, lisible, efficace efficace pour soutenir la rémunération des salariés et des indépendants qui travaillent dans des conditions délicates et assurent la continuité de la vie économique. C'est pour nous, aussi, essentiel. Il faudra informer le Parlement, de manière précise et régulière, sur le déploiement des mesures de soutien à l'activité économique, ainsi que sur l'impact de la crise sur l'hôpital public et les collectivités locales. Le second courrier souligne l'engagement pris par le Gouvernement, dimanche, en séance publique- par votre voix, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement -, d'informer mensuellement les commissions permanentes du Sénat des mesures prises en application de la loi d'urgence destinée à faire face à l'épidémie de Covid-19. Cette information porte sur trois points les actes pris par l'exécutif et ses représentants locaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; les dispositions envisagées par le Gouvernement dans les ordonnances et leurs décrets d'application-

des ministres ; les mesures prises pour assurer la continuité du fonctionnement des assemblées délibérantes locales et les modalités d'organisation du second tour des élections municipales. Le Sénat entend accomplir la plénitude des missions confiées à ses soins par la Constitution, dans le respect des contraintes que nous impose la situation sanitaire et dans un juste équilibre entre ces contraintes et l'exigence démocratique. Je sais pouvoir compter sur vous, monsieur le Premier ministre, pour établir entre nous une collaboration confiante, et le Gouvernement sait pouvoir compter sur le Sénat. Je souhaite également qu'une attention toute particulière soit portée à nos compatriotes des outre-mer

chers collègues, que nous ferons nôtre la priorité sanitaire. Notre séance de questions est, comme à l'accoutumée, retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

d'abord, la rumeur sur la participation des hôpitaux privés est inexacte. L'ensemble des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, se sont vu intimer la consigne très stricte d'arrêter toute activité programmée depuis plusieurs semaines déjà et de libérer toutes les places en soins intensifs et en réanimation.

et des Ehpad, notamment dans les régions où le virus circule le plus. Je n'ai pas caché la situation. La consommation de masques est encore plus massive du fait des caractéristiques du virus. Dans les territoires et hôpitaux dans lesquels il circule, il est fondamental de protéger prioritairement les personnes travaillant dans les services de réanimation auprès des malades les plus graves. C'est indispensable ! J'ai autorisé, comme le Haut Conseil de la santé publique le demandait, la prescription collégiale,

La situation est compliquée, monsieur le ministre. Je comprends que vous écoutiez les remontées de votre administration- c'est tout à fait légitime -, mais écoutez aussi les remontées des élus : la grogne est en train de la grogne est en train de monter ! Peut-être qu'en période de guerre on pourrait prendre des décisions qui ne soient pas scientifiquement correctes, mais qui permettraient parfois de soigner la population

Hier, les marchés ont été interdits, dans des conditions qui peuvent d'ailleurs faire débat. Pour compenser le manque à gagner, le ministre de l'économie a enjoint la grande distribution- on peut être d'accord avec lui sur ce point -à acheter des produits français.

lorsqu'ils sont sans activité, ils aillent travailler dans les champs. Cette déclaration a d'abord suscité l'incompréhension : alors que les mesures de confinement viennent d'être renforcées, comment des centaines de milliers de personnes pourraient-elles rejoindre les campagnes pour prêter main-forte aux agriculteurs ? ? Pourtant, l'appel semble avoir été entendu, puisque plus de 40 000 personnes se seraient déjà portées volontaires. Hier soir, tard, le Gouvernement a annoncé par communiqué la création d'une plateforme dédiée. lors, plusieurs questions se posent : comment ce dispositif va-t-il fonctionner, en particulier dans quelles conditions sanitaires ? Si la mobilisation est insuffisante, comment notre agriculture pourra-t-elle continuer de répondre à la demande ? N'y a-t-il pas un risque de pénurie ? Ce sont des questions légitimes que se posent nos agriculteurs et les Français. La parole est à Mme la ministre du travail. Oui, monsieur

La République En Marche. Monsieur le ministre des solidarités et de la santé, depuis lundi minuit, les vols entre l'Hexagone et l'outre-mer sont interdits, sauf dérogations exceptionnelles. Les outre-mer ne sont pas épargnés par cette pandémie plus de 330 cas confirmés de coronavirus sont à ce jour diagnostiqués, qui s'ajoutent parfois, comme c'est le cas à Mayotte et à La Réunion, à ceux liés à l'épidémie de dengue, d'une exceptionnelle ampleur. Ce nombre est certainement sous-estimé. apparence moins touchés, leur situation sanitaire compliquée, liée à leur insularité, leur isolement et leur éloignement, mais surtout à la faible capacité d'accueil des malades, fait unanimement craindre une explosion du nombre de contaminations. Mon département, qui a connu son premier cas le 14 mars, en compte aujourd'hui trente-cinq. Vous connaissez la faiblesse du système de santé à Mayotte. Malgré le travail considérable des professionnels soignants, que je tiens ici à remercier chaleureusement, l'hôpital, déjà saturé, ne compte que seize lits de réanimation et seuls vingt-huit médecins libéraux exercent sur ce territoire, pour une population officielle de 257 000 habitants, mais qui s'élève probablement au double en raison de l'immigration clandestine. Une grande partie de la population vit dans des conditions de précarité et de promiscuité propices à l'expansion de cette épidémie. Sur place, les gestes barrières et de confinement ne sont pas bien respectés, souvent par impossibilité. Comment faire autrement lorsque l'on vit à plusieurs dans une habitation traditionnelle sans accès aux sanitaires ? Mais à ceux qui peuvent respecter ces règles et qui agissent par insouciance, je le redis : ne prenez pas ce virus à la légère, ne croyez pas que le climat ralentira sa progression et restez chez vous pour protéger vos familles Hier, par audioconférence, le préfet et les élus de Mayotte, tous très mobilisés, ont fait le point. Monsieur le ministre, hormis les mesures sur les transports aériens, pourriez-vous nous dire quelles sont les dispositions prises par le Gouvernement pour aider les territoires ultramarins, particulièrement vulnérables, à faire face à cette pandémie ?

C'est la raison pour laquelle nous avons pris des décisions, très rudes, de limitation, voire de très grande limitation, des vols commerciaux à destination des outre-mer, afin de limiter au maximum

C'est pourquoi aussi, en plus des restrictions portant sur l'utilisation des vols commerciaux, nous avons imposé à tous ceux qui partaient vers les territoires ultramarins une quatorzaine stricte à leur arrivée. Néanmoins, vous savez comme moi qu'un certain nombre de cas sont à déplorer en Guadeloupe, à la Martinique,

Le 23 mars dernier, la décision est tombée comme un coup de massue sur les territoires : le Gouvernement a interdit l'ensemble des marchés, sauf autorisation du préfet accordée après avis du maire. Pourtant, sur le terrain, de nombreux marchés avaient déjà mis en place de bonnes pratiques allant bien au-delà de celles des grandes surfaces, dans lesquelles les clients peuvent circuler et manipuler librement les produits. Pourquoi créer du gaspillage alimentaire ainsi qu'une rupture d'égalité de traitement entre les grandes surfaces et les marchés, où se trouvent des acteurs locaux porteurs de résilience ? ? Par cette décision, en effet, ce sont notamment des petits producteurs en vente directe, mais aussi des acteurs de la pêche artisanale et des ostréiculteurs qui voient leur survie économique menacée. Alors que l'alimentation est un secteur stratégique, n'est-il pas nécessaire de soutenir et de sécuriser les marchés et l'ensemble des initiatives de vente directe ?

Oui, il faut faire confiance aux maires ! Mais se sentiront-ils en confiance pour demander des dérogations, alors que les préfets ont des interprétations diverses de l'arrêté et que certains ont déjà refusé des demandes ? avoir une parole bien claire pour encourager les maires et les préfets à maintenir les marchés et les pratiques de vente directe dans le respect des règles sanitaires ? La parole est à M. le Premier ministre.

Ces dérogations doivent être accordées par les préfets, après demande et avis des maires, lesquels sont mieux placés que quiconque pour apprécier si, dans telle commune,

L'heure est grave. L'épidémie de coronavirus s'étend sur toute la planète, et notre pays est particulièrement frappé. Des mesures exceptionnelles sont prises, mais elles ne sont pas suffisantes. Nos hôpitaux, nos Ehpad appellent

est dramatique. Cette incapacité est révélatrice du ravage du libéralisme, système que vous portiez aux nues avec d'autres- mais ça, c'était avant ... L'État doit maintenant reprendre la main, un État citoyen au service du peuple.

seul fabricant en Europe de bouteilles d'oxygène, usine fermée il y a quinze mois par son propriétaire britannique. Les 134 ex-salariés ont maintenu en état le matériel. Annoncez la nationalisation et la réouverture réouverture ! Il faut réquisitionner des usines de textile pour la fabrication massive de masques. Contrairement à d'autres, elles sont aujourd'hui indispensables à la gestion de l'urgence sanitaire. Oui, Emmanuel Macron a raison quand il déclare qu'un modèle de développement dévoile ses failles au grand jour

construites sur la quête du profit, la concurrence, la primauté des intérêts privés vacillent. La crise sanitaire en est le terrible révélateur. Oui, il faut redonner à l'État la maîtrise du destin de notre pays ! Mais, contrairement au Medef, nous ne voulons pas de nationalisations temporaires

auxquels s'ajoutent 300 milliards de garanties apportées par l'État sur les prêts consentis par les banques. Il ne s'agit pas de défendre les banques, il s'agit de faire en sorte que les entreprises puissent obtenir un financement pour continuer à vivre

cet effort de redémarrage sera certainement considérable. Il ne devra d'ailleurs pas être seulement national, même s'il aura évidemment une dimension nationale ; il devra aussi être coordonné aux niveaux européen et mondial. Bref, il y aura un champ considérable d'actions économiques collectives et publiques à mettre en oeuvre. Vous avez évoqué l'instrument des nationalisations. L'État est d'ores et déjà actionnaire d'un certain nombre de grands groupes qui lui paraissent stratégiques ou pour des raisons historiques, les deux n'étant pas incompatibles.

intervenir- au-delà des entreprises dans lesquelles l'État est déjà actionnaire -soit par des prêts particuliers, soit par des prises de participation dans des entreprises que nous jugeons stratégiques

pour déterminer où et quand il conviendra d'intervenir en fonction de la capacité desdites entreprises à passer cette période délicate et de leur caractère stratégique ou non pour le tissu productif national ou pour la souveraineté française. Je vous ai répondu de manière générale, j'en ai conscience,

Je souhaite avant tout avoir une pensée pour tous nos concitoyens, qu'ils soient confinés chez eux, touchés par la maladie, par le deuil, mais aussi pour l'ensemble de nos compatriotes qui assurent en ces jours des fonctions essentielles et vitales au en termes de santé, d'entretien, d'alimentation, de sécurité, d'enseignement, de production ou encore de continuité du service public. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le Gouvernement, le Parlement et les collectivités ont dû adopter des mesures sanitaires strictes, mais vitales. Alors que la période de confinement initialement annoncée sera prolongée, nous pouvons constater de premières conséquences économiques et sociales. Je pense à la tension naissante sur certains prix déjà visible dans l'Hexagone et dans les outre-mer. Il nous incombe donc d'être préparés dès à présent aux conséquences de la crise sur le pouvoir d'achat des Français. Nous devons anticiper cette situation et prendre des décisions immédiatement.

Nous demandons également au Gouvernement de mettre en place un dispositif pour maintenir le pouvoir d'achat des agriculteurs et des producteurs. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire quand sera pris ce décret de blocage temporaire des prix ?

Monsieur le Premier ministre, dans une crise sanitaire, comme dans toute catastrophe, l'action publique doit d'abord parer au plus urgent : protéger les vies humaines, quoi qu'il en coûte. C'est la ligne retenue par le Gouvernement, celle aussi soutenue par le Parlement et surtout celle attendue par les Français. Pour commencer, je voudrais donc me joindre à l'hommage rendu par les orateurs qui m'ont précédé à tous les personnels soignants de notre pays. en oeuvre des mesures drastiques pour limiter l'expansion du virus, il faut agir avec autant de force pour que l'économie ne s'effondre pas. Nous y avons contribué en adoptant dimanche dernier les deux projets de loi que vous nous aviez soumis. Le Gouvernement dispose désormais d'importants moyens pour tendre à nos entreprises de nécessaires filets de sécurité. Mais l'État ne peut pas tout. Alors que tout indique un ralentissement globalisé de l'économie, la mobilisation du secteur privé sera également indispensable aucune des forces vives du pays ne doit manquer à l'appel. Bon nombre de nos entreprises accusent le coup et s'apprêtent à ouvrir des lignes de crédits garantis par l'État. l'État. Pour remettre les entreprises sur les rails de l'activité, l'action des professionnels de l'assurance sera également nécessaire. La couverture d'un risque consiste pour l'essentiel à évaluer la probabilité qu'un événement se produise, ainsi que les dégâts financiers qu'il pourrait causer. Lorsque l'événement est inédit et les dégâts incommensurables, la tâche évidemment se complique ... De très nombreuses entreprises font savoir que les pertes d'exploitation qu'elles subissent actuellement ne sont pas couvertes par leurs contrats d'assurance. Leurs dirigeants sont bien sûr très inquiets. Monsieur le Premier ministre, que peut faire le Gouvernement pour adapter le cadre assurantiel à la gravité de la situation que nous connaissons ? L'état d'urgence sanitaire qui vient d'être institué a-t-il vocation à intégrer un volet assurantiel, par exemple sur le modèle du régime existant en matière de catastrophes naturelles ?

ne fais pas de fétichisme du chiffre, mais vingt-cinq est un nombre considérable. Ces ordonnances permettent, secteur par secteur et sujet par sujet, d'essayer d'apporter des solutions juridiques

aux pertes qui résulteraient d'une cause autre qu'un dommage matériel. Autrement dit, les contrats actuels n'ont pas, pour l'immense majorité d'entre eux, prévu ce type de dommage, d'accident, d'aléa.

aux toutes petites entreprises qui se trouvent confrontés à l'interruption de leur activité. Le deuxième élément utile est le maintien des garanties d'assurance des TPE qui connaîtraient des difficultés ou des retards de paiement pendant toute la durée de la période de suspension de l'activité. Cela dès lors qu'il n'y a pas de recettes, il ne pourra pas y avoir de perte de droits parce qu'il n'y aurait plus de paiement des polices d'assurance. Cet engagement important a été pris par le secteur, et il sera garanti. Enfin, même s'il est probablement trop tôt pour tirer tous les enseignements de cette crise mais il sera utile d'y réfléchir très rapidement, le ministère de l'économie et des finances

aux TPE, commerçants et artisans qui vont rester ouverts parce que leur activité est considérée comme essentielle, mais qui subiront tout de même une perte de chiffre d'affaires. Il faudrait les aider : êtes-vous prêt à agir en ce Le dispositif des 1 500 euros pour ceux qui ont perdu 70 % de leur chiffre d'affaires par rapport à mars 2019 sera de peu d'effet. Le report des charges ou des factures de gaz ou d'électricité à quelques mois

D'abord, je voudrais relever les points positifs. Je vous remercie de souligner que la garantie d'emprunt apportée par l'État, à hauteur de 300 milliards d'euros, est un élément favorable qui doit évidemment être mis en oeuvre avec le soutien des banques. J'ai cru comprendre, à la lecture d'un certain nombre de messages ce matin, que les banques, la fois, le vote favorable du Sénat que vous avez mentionné et la promulgation de la loi, avaient déjà commencé à faire part à leurs clients de leur disponibilité à accorder ces emprunts. Je sais que certaines banques ont été très réactives. Notre objectif est évidemment que cet instrument serve, les entreprises en ont besoin. Je ne méconnais pas les difficultés qui, çà et là, peuvent se poser compte tenu du plan de charges des agences ou de la difficulté à faire en sorte que l'ensemble de celles-ci fonctionnent dans de bonnes conditions. Mais je peux vous faire état, monsieur le sénateur, de la grande mobilisation du secteur bancaire et de la volonté que cet instrument puisse porter tous ses fruits.

dans notre dispositif, les entreprises ne subissent aucune perte si elles décident de passer en chômage partiel et les salariés voient leur revenu garanti à une hauteur qui est supérieure à ce qui se fait dans d'autres pays, y compris l'Allemagne.

les commandes sont passées, les avions sont affrétés et ils devraient servir dans des délais très brefs. Croyez-moi, je suis le premier à faire en sorte que cela se passe ainsi, puisque nous avons besoin de cette ressource. Je pense que tout se passera correctement, mais permettez-moi, monsieur le sénateur,

Je m'associe aux hommages que vous avez formulés, mes chers collègues, à l'endroit de nos concitoyens qui travaillent dans des conditions très difficiles, au premier rang desquels les personnels de santé, mais aussi les professionnels de tous les secteurs qui permettent aux Français de disposer des biens et services indispensables. Je souligne également l'investissement des fonctionnaires de nos services publics, dont on réalise, plus encore en ces périodes de crise majeure, qu'ils sont, non pas une dépense, mais un investissement, une protection dont on ne peut se passer. Les maires et les élus locaux sont également en première ligne. L'unité nationale ne doit pas empêcher le débat démocratique, et je veux me faire la porte-parole des interrogations exprimées par nos concitoyens sur les mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Le renforcement du confinement protège et sauve des vies, mais il est grand temps de mettre tout en oeuvre pour se doter de masques, de tests de dépistage, de gels hydroalcooliques, de respirateurs, qui continuent de manquer scandaleusement. Quand les personnels mobilisés pour combattre cette épidémie disposeront-ils de ces éléments de protection et de soins élémentaires ? Il faut tirer les leçons de cette crise sanitaire sans précédent et, dès maintenant, augmenter les moyens financiers et humains qui manquent cruellement à notre système de santé. santé) demande la généralisation des tests de dépistage du Covid-19 afin de confiner les personnes positives et, ainsi, éviter de nouvelles contaminations. Les tests disponibles à ce jour et dans les jours qui viennent seront absolument insuffisants, notamment au regard des 800 000 résidents des Ehpad menacés d'une effroyable hécatombe si des dispositions drastiques ne sont pas prises de toute urgence. Monsieur le ministre, quand vous rangerez-vous à ces recommandations de l'OMS et quand ces tests seront-ils enfin généralisés dans notre pays ?

sur les annonces que j'ai faites. Nous allons continuer de nous conformer scrupuleusement aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de tests. Les recommandations ont évolué avec la connaissance du virus, les recommandations ont évolué avec l'apparition de la pandémie, les recommandations ont évolué avec l'identification des différentes stratégies mises en place dans tous les pays qui ont fait face en même temps que nous, ou quasiment en même temps que nous, à l'épidémie. Ces pays ont choisi des

à déconfiner la France, à l'heure où les Français seront amenés à quitter leur domicile pour retrouver une vie normale. L'enjeu de ces tests sera surtout de savoir qui aura été malade et qui ne l'aura pas été.

pour le groupe Union Centriste. La fermeture des écoles et établissements scolaires a plongé l'ensemble du système éducatif dans une situation inédite. Dans ces conditions difficiles, je tiens à saluer l'implication des directeurs d'établissement et des enseignants, qui assurent la continuité pédagogique et le respect des programmes dans notre pays. Si le constat est globalement positif, quelques questions

De surcroît, le rôle des parents est essentiel et pallie l'absence contrainte des enseignants. Il existe de grandes disparités entre les familles au sein desquelles les parents sont disponibles pour aider tout au long de la journée leur enfant et celles où les parents sont nécessairement moins présents. Le risque est grand de voir une forme de décalage se renforcer entre deux catégories de familles : celles qui disposent du temps nécessaire, de la maîtrise des derniers outils technologiques et les autres. La question du rattrapage, une fois le confinement terminé, se posera pour certains enfants. Les familles sont en demande d'information de la part des enseignants sur le rôle qu'elles doivent tenir dans l'accompagnement pédagogique des enfants. Il semblerait qu'il existe des disparités

dans quelques jours, des maires pourraient recevoir des courriers leur indiquant la fermeture de classes dans leurs écoles. Dans la période actuelle, il apparaît opportun de suspendre ce calendrier et d'éviter des tensions supplémentaires dont nous n'avons pas besoin. Par ailleurs,

Avant de conclure notre séance, je vous rappelle, mes chers collègues, que le droit de questionnement continue également à s'exercer sous la forme des questions écrites